cohérent de considérer qu’elles n’ont pas vocation à faire usage de ces dispositifs d’hébergement, lesquels sont saturés. Le présent amendement tend à s’inscrire en cohérence avec le vote par le Sénat d’une disposition comparable concernant les déboutés du droit d’asile,

telle inclusion des places d’hébergement dans le décompte de la loi SRU, vieille lune de la droite sénatoriale, est fallacieuse, puisqu’elle va permettre à certaines communes de s’exonérer de la construction de logements sociaux au motif que des centres d’accueil se trouvent sur leur territoire. En effet, faire entrer dans le domaine des logements sociaux ces centres d’hébergement temporaire leur permettrait de simuler un effort de contribution à la construction de logements sociaux et d’éviter ainsi toute sanction financière. Ils pourraient alors préserver un égoïsme social contraire au pacte républicain, à la solidarité territoriale à la nécessaire mixité sociale qui en découle. En République, il n’y a pas à choisir entre des logements sociaux et des structures d’hébergement temporaire. Il ne nous semble donc absolument pas opportun que certaines collectivités prennent prétexte de cette exigence d’humanité qu’est l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés pour s’exonérer de leur obligation de construction de logements sociaux. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Quel

L’instauration d’une procédure d’éviction du lieu d’hébergement des personnes nouvellement reconnues comme réfugiées, aujourd’hui restreinte aux personnes déboutées, mettrait sérieusement en péril leur intégration en France. Elle provoquerait leur mise à la rue et les priverait de l’accompagnement dont elles bénéficient. Ce projet de loi supprime le délai d’un mois, qui permettrait aux personnes de prendre leurs dispositions pour quitter leur lieu d’hébergement, en les obligeant à en sortir immédiatement après la décision de la CNDA, sauf décision du préfet. Cette disposition n’est pas conforme au droit européen et risque de mettre dans un dénuement extrême encore plus de demandeurs d’asile. L’inconditionnalité de l’accueil doit être défendue et respectée comme un principe intangible

telle possibilité existe déjà dans le droit, elle est à la discrétion de l’administration. Il n’est donc pas nécessaire de l’inscrire dans la loi. En outre, une telle décision pourrait avoir des conséquences dommageables pour les personnes les plus vulnérables. Une femme enceinte pourrait, par exemple, se retrouver à la rue.

l’autorité préfectorale a parfaitement la possibilité de ne pas prendre cette décision et d’y déroger. Ce dispositif me paraît équilibré.

s’il a présenté une demande de réexamen ou si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité ou la sûreté de l’État. L’intérêt supérieur du mineur exige un examen bénéficiant de

Ainsi, sur les 44 mesures du dernier plan d’action national contre la traite des êtres humains, seulement 3 ont été mis en œuvre : 3 sur 44 ! Il est temps de renforcer cette lutte. Les dispositions de cet amendement se veulent un pas concret vers une meilleure protection des victimes de la traite dès lors que celles ci parviennent à s’en extraire. On le sait, il est extrêmement difficile de sortir de l’emprise des organisateurs de la traite, qui confisquent toute pièce d’identité et menacent la personne avec des mesures de rétorsion très graves, comme l’assassinat de proches, dès lors que la victime tente de s’extraire de la traite. Quelques victimes y parviennent tout de même ou sont libérées à la suite du démantèlement d’un réseau. Quand elles réussissent, nous leur devons une protection. Or cette protection n’est pas garantie aujourd’hui pour les victimes de la traite qui déposent une demande d’asile une fois qu’elles car cette demande peut tout simplement être traitée en procédure accélérée. C’est totalement inapproprié, puisque cela ne permet pas d’examiner la demande en détail et limite le droit au recours de la victime contre une décision de refus. Étant donné que les réseaux de la traite s’étendent souvent entre une multitude de pays et qu’ils se caractérisent par leur complexité, les parcours des victimes, eux aussi, s’étendent souvent sur plusieurs pays. Or la demande peut être examinée en procédure accélérée pour le motif que le pays d’origine est considérée comme « sûr ». Ce classement revient, de fait, à méconnaître entièrement les horribles réalités des réseaux de la traite, d’où l’intérêt de cet amendement.

l’article 20 fait partie du titre IV, « Engager une réforme structurelle du système

assurer une qualité d’écoute, comprendre les situations politiques pointues des pays d’origine

bien. Le cœur du projet du Gouvernement, indépendamment de la lutte contre les délinquants étrangers et de l’exigence d’intégration, est donc la simplification des procédures au sens très large du terme, notamment des procédures d’asile, qui connaissent un détournement.

Comme le soulignent de nombreuses associations, depuis 1952, la Commission des recours des réfugiés, puis la CNDA, qui lui a succédé, est une juridiction collégiale composée d’un magistrat administratif et quelquefois d’un magistrat judiciaire, ainsi que de personnalités qualifiées nommées par le vice président du Conseil d’État et surtout par le Haut Commissariat aux réfugiés. Cette spécificité est à nos yeux gage d’impartialité. Or c’est ce que l’article 20 propose de supprimer, au nom d’une prétendue efficacité. Certes, il est nécessaire

Or, comme le soulignent de nombreuses associations, la présence de trois juges permet de croiser les regards et d’éviter de se laisser guider par des représentations personnelles pour juger de la crédibilité et la cohérence du récit de la personne demandant refuge et asile. Selon Amnesty International, « Une journée d’audience, ce sont treize dossiers examinés, treize histoires de vie très différentes : d’un opposant politique sri lankais à une jeune fille fuyant l’excision en Guinée, en passant par des persécutions liées à l’orientation sexuelle… Trois juges ne sont pas de trop lorsqu’il s’agit de traiter de dossiers si sensibles. De nombreuses personnes qui demandent l’asile jouent leur vie et leur sécurité à ces audiences. » C’est pourquoi nous nous opposons à toutes les mesures visant à amoindrir les garanties offertes aux demandeurs d’asile, en particulier dans des audiences où l’intime conviction est le principal critère de décision.

lorsqu’il examine la conformité d’une loi aux normes constitutionnelles. De même, le Conseil d’État a reconnu « la particulière importance que revêt, pour les demandeurs d’asile, la garantie d’un examen de leur recours par une formation collégiale, telle qu’instituée en principe par le législateur

Les affaires jugées à la CNDA étant très complexes, elles doivent donner lieu à ces échanges, en particulier lors des audiences, compte tenu de la forte dimension orale du contentieux de l’asile.

de ce magistrat de la CNDA qui a été écarté de ses fonctions en raison de ses publications sur les réseaux sociaux. Pour éviter ces écueils, cet amendement a pour objet de ne pas revenir sur le principe de la collégialité comme procédure ordinaire. L’amendement

peut renvoyer devant une formation collégiale « s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie ».

dans le cadre de la formation continue, la CNDA organise trois formations par an sur les mêmes thématiques, pour une durée de trente cinq heures chacune, ce qui ne me paraît pas négligeable.

le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin ne décide, à tout moment de la procédure, d’inscrire l’affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.

sur l’initiative de ma collègue Mélanie Vogel, propose d’élargir l’évaluation de la vulnérabilité des demandeuses d’asile aux victimes d’agressions sexuelles. Les femmes qui demandent l’asile en France

témoignent régulièrement de violences faites aux femmes, dont des mariages forcés, des violences conjugales et des mutilations sexuelles, y compris envers les filles de la demandeuse. En second lieu, les violences commises dans le pays d’origine sont malheureusement loin d’être les seules auxquelles s’exposent les demandeuses d’asile.

ONU Femmes alerte sur le fait que les femmes et les enfants deviennent souvent victimes d’agressions sexuelles lors de leur parcours migratoire, et ce non seulement une fois, mais à plusieurs reprises. Ainsi, sur la route migratoire entre la Libye et l’Italie,

Cette situation gravissime, vécue quotidiennement par les personnes étrangères, découle directement de la dématérialisation des prises de rendez vous,

pour obtenir des rendez vous en préfecture, en raison de l’absence de créneau disponible sur internet. Les tribunaux administratifs nous expliquent même qu’ils sont devenus les secrétariats des préfectures… Dans sa décision du 27 novembre 2019, le Conseil d’État concluait qu’une solution de rechange à la saisine par voie électronique devait toujours être proposée. Tel n’est pas le cas aujourd’hui. Le manque de personnel en préfecture pour traiter les dossiers, la dématérialisation et la disparité des pratiques préfectorales ne font qu’allonger les délais d’attente pour obtenir une régularisation ou le statut de réfugié. Le GEST encourage le Gouvernement à transformer l’essai et à financer les services de préfecture à la hauteur des enjeux qu’ils traitent, notamment pour les étrangers. Nous aurons l’occasion d’en discuter dans le cadre du projet de loi de finances, puisque nous ne pouvons pas le faire

Le dysfonctionnement du service d’accueil des étrangers en préfecture est tel que certains sont en effet contraints de demeurer en situation irrégulière, au risque d’être expulsés du territoire. Pour les personnes voulant demander le renouvellement de leur droit au séjour, séjour, l’impossibilité d’accéder aux services de la préfecture peut entraîner des ruptures ou un non renouvellement des contrats de travail, ainsi qu’une interruption de l’assurance maladie ou du versement des prestations sociales. La vie des gens tient donc au fonctionnement kafkaïen, disons le, des services d’accueil des étrangers.

La situation est d’autant plus alarmante qu’elle entraîne ensuite un engorgement des tribunaux administratifs, le recours contentieux devenant un préalable presque obligatoire à l’accès aux guichets préfectoraux. Ce n’est pas acceptable, ni pour les usagers ni d’ailleurs pour les agents, qui sont placés dans des situations épouvantables, que ce soit dans les collectivités, les tribunaux ou les préfectures. La volonté de contrôler les flux migratoires ne saurait passer par une détérioration insidieuse des conditions insidieuse des conditions d’accueil des usagers et de travail des agents. Les ressortissants étrangers qui se présentent en préfecture, quelle que soit leur situation administrative, sont des usagers. À ce titre, ils sont dignes de respect. C’est le sens de notre demande de rapport sur l’impossible accès des personnes étrangères en préfecture et sur les mesures envisagées pour y remédier. Quel est l’avis la commission ? Ces deux amendements

% ! Ce dernier est devenu le premier motif de saisine de l’institution, passant de 10 % à 24 % des réclamations reçues par l’institution. Cet accroissement concerne essentiellement l’obtention de rendez vous, les difficultés en lien avec la dématérialisation des guichets et les délais d’instruction excessifs. Par cet amendement, nous proposons au Gouvernement, d’une manière qui est certes détournée, mais qui est la seule que nous puissions utiliser dans le cadre de ce projet de loi,

sur lequel nous devons fonder toute notre réflexion et mobiliser les moyens de la justice est celui de la restriction des libertés. Le délai de soixante douze heures applicable dès lors que la mesure d’éloignement n’est pas assortie d’un départ volontaire, quand bien même l’étranger ne serait pas retenu,

le week end. En cas de placement en rétention, le délai bref se justifiait par la privation de liberté et la présence d’associations dans les centres de rétention, qui permettent à l’étranger un premier accès au droit effectif et la défense de ses droits.

une bonne idée. Il introduit une de recours applicable à l’ensemble des obligations de quitter le territoire français et aux actes administratifs qui y sont liés. Le délai de recours laissé au requérant est de trente jours. Le tribunal administratif statue en formation collégiale, en principe dans un délai de six mois. Cette

En effet, le projet de loi prévoit un recours dérogatoire urgent pour les OQTF prononcées sans délai de départ volontaire, le requérant ayant soixante douze heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en juge unique dans un délai de six semaines. il est très difficile pour un requérant de trouver un conseil en soixante douze heures. Le Conseil d’État recommande de ne réserver une procédure d’urgence que lorsque cela est justifié par une mise à exécution forcée de l’éloignement, c’est à dire en cas de placement en rétention.

La pratique administrative favorise la prise d’OQTF sans délai de départ volontaire, mais ne l’assortit que rarement d’un placement en rétention immédiat qui justifierait le recours à une procédure contentieuse d’urgence. Il est donc injustifié

prévoit la tenue de l’audience, par principe, dans une salle délocalisée aménagée à proximité du lieu d’enfermement. De plus, sur décision du magistrat, cette audience peut se tenir en visioconférence.

Ces méthodes ont pour effet de chasser le retenu du tribunal. Dès lors que le juge administratif peut choisir de se rendre dans la salle d’audience délocalisée ou de tenir audience au tribunal, le Conseil d’État, dans son avis, estime que « ces dispositions induiront un recours accru à la visio audience ». Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le Conseil d’État ! Ces nouvelles modalités de jugement inhumaines et discriminantes sont, selon le Conseil national des barreaux, contraires au droit au procès équitable, qui suppose l’accès au juge, la publicité de l’audience et une égalité des armes. La visio audience prive les justiciables d’une défense effective, s’agissant du contentieux de l’urgence de personnes vulnérables. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’oppose fermement à la dématérialisation des audiences, pour des raisons liées à l’exigence de solennité de ces dernières, défendre le respect du contradictoire. Je précise que cet amendement a été travaillé à partir des propositions de l’Union syndicale des magistrats

reste la tenue de l’audience dans les locaux du tribunal administratif compétent, afin que la visioconférence soit réservée aux seuls cas de force majeure, tel un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant. À défaut, elle devrait être conditionnée à l’accord préalable du requérant.

Le projet de loi prévoit la possibilité de recourir aux visio audiences, afin de simplifier le déroulement des audiences pour le contentieux des étrangers. Nous comprenons bien entendu l’objectif de simplification, mais il ne saurait à lui seul justifier des transgressions excessives par rapport au respect des droits des justiciables. Hélas, nous observons cette tendance au renoncement depuis quelques années. Et la crise du covid 19 n’a pas aidé à la freiner. Par cet amendement, nous nous associons à la Défenseure des droits, qui, dans son avis du 23 février a souligné que ces mécanismes ne permettaient pas « de garantir la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ni d’assurer la confidentialité de la transmission ». Nous proposons donc de revenir sur cette possibilité en limitant à deux cas de figure le déroulement de l’audience : dans une salle aménagée du CRA ou dans les locaux du tribunal administratif compétent.

acteurs – le juge, le greffier, l’étranger, l’avocat et l’interprète – et met à mal le principe de publicité des débats, garant d’une justice de qualité, en raison de l’éloignement géographique de ce lieu de justice : il nous paraît nécessaire d’offrir aux magistrats la faculté de décider souverainement si l’audience peut être délocalisée sans porter atteinte à la publicité et au bon déroulement des débats. Cet amendement tend donc à ajouter une dérogation si les magistrats constatent que les conditions d’accès à la salle ou au lieu où elle se situe ne permettent pas d’assurer effectivement cette publicité des débats. Je vous remercie

que cette remise en cause du caractère suspensif du recours porte atteinte au principe d’égalité de traitement des recours et au droit à un recours effectif des demandeurs d’asile, dans la mesure où elle permet l’éloignement d’un étranger, alors même que son recours est toujours pendant devant la CNDA. Certes, le Conseil constitutionnel a validé cette remise en cause, mais au prix d’une véritable usine à gaz : on demande au tribunal administratif de se prononcer sur la possibilité du demandeur de rester sur le territoire, alors même que la procédure de demande d’asile n’est pas terminée.

le recours n’est pas suspensif ne privait pas l’intéressé de son droit à un recours effectif. Nous ne voyons pas de raison d’aller au delà de l’appréciation du juge constitutionnel.

pour la sécurité de nos concitoyens. Quand nous signons un arrêté ministériel d’expulsion, nous devons, en vertu du code de justice administrative, partager avec la partie adverse l’intégralité de nos informations. Or il

lors de l’instruction d’un litige lié au refus d’un titre de séjour « étranger malade », cet article porte atteinte à une obligation déontologique majeure, à un droit fondamental. Encore une fois, les droits les plus élémentaires des personnes étrangères sont bafoués au nom d’une obsession migratoire, alors même que plusieurs textes législatifs et réglementaires propres au droit du séjour et à la protection contre l’expulsion des personnes étrangères malades rappellent l’importance de la préservation du secret médical par rapport à l’autorité administrative et le choix laissé à la personne concernée d’une éventuelle levée de ce secret. Restreindre ainsi ce droit fondamental,

les patients de recourir à des soins médicaux essentiels, par crainte que leurs informations médicales ne soient utilisées contre eux dans des procédures administratives. Cela pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour la santé publique, en retardant le diagnostic et le traitement de certaines en particulier pour les personnes vulnérables. Le droit au secret médical est un pilier de l’éthique médicale. Le serment d’Hippocrate dispose : « Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. » les professionnels de santé sont tenus de protéger les informations médicales de leurs patients, et cela ne doit pas être compromis par des considérations administratives. L’atteinte au secret médical est une mesure d’exception, qui ne devrait être autorisée que dans des circonstances strictement définies par la loi et en respectant les droits des individus concernés, c’est à dire leur consentement. Quel

ou à son délégué de déclarer son recours suspensif, lorsqu’il lui semble que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation ou en cas de menace grave pour l’ordre public.

Selon le Syndicat de la juridiction administrative (SJA), la justice administrative doit être rendue dans des lieux particuliers, identifiés et identifiables comme lieux de justice, afin de préserver et de garantir la force symbolique de l’audience et de la décision de justice.

La généralisation de ce dispositif représente une justice bâclée, rendue dans des conditions déshumanisantes. La justice ne doit pas être rendue dans un lieu autre qu’un lieu de justice – c’est une garantie offerte par notre République –, notamment dans un local annexe d’un centre de rétention administrative ou d’un aéroport, fût il baptisé « salle d’audience », pour des raisons liées à l’exigence de solennité, mais aussi à des considérations techniques et pratiques. Les étrangers doivent pouvoir bénéficier par exemple du soutien de leurs proches ou de leur famille. L’exigence d’impartialité objective impose aussi que les contentieux mettant en cause les services du ministre de l’intérieur

délocalisée sans porter atteinte à la publicité et au bon déroulement des débats. Cet amendement tend donc à ajouter une dérogation si les magistrats constatent que les conditions d’accès à la salle ou au lieu où elle se situe ne permettent pas d’assurer effectivement cette publicité des débats.

La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a modifié la condition liée au consentement de la personne pour la tenue des audiences en vidéoconférence, alors que le dispositif porte une atteinte forte au droit à la défense de la personne intéressée. Selon le rapport de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers, l’usage de la visioconférence transforme radicalement le déroulement de l’audience. Même lorsque le dispositif relie deux salles d’audience censées présenter les mêmes garanties, la personne étrangère qui comparaît par visioconférence voit […] son droit à un procès équitable sérieusement mis à mal. La procédure contradictoire implique notamment que la personne étrangère puisse comprendre les arguments avancés et présenter ses observations. Elle implique également le droit de s’entretenir dans de bonnes conditions avec son avocat. Si la personne étrangère est physiquement mise à distance par le biais de la visioconférence. Elle n’a presque plus aucune chance ni de comprendre ce qui se passe dans la salle d’audience du côté du juge ni de réussir à s’exprimer utilement. La présence en un même lieu du juge, du justiciable et de son conseil, c’est à dire le face à face judiciaire, est absolument nécessaire pour que la personne étrangère comprenne les enjeux attachés à l’audience et à la décision judiciaire qui en résulte.

du préfet. Le Conseil constitutionnel a rappelé dans une décision du 25 février 1992 que « le maintien d’un étranger en zone de transit, en raison de l’effet conjugué du degré de contrainte qu’il revêt et de sa durée,

d’incapacité des services du ministère de la justice. Il pèsera pourtant sur les étrangers. Les zones d’attente sont des lieux privatifs de liberté très anxiogènes, où les personnes sont contraintes et surveillées. Parmi elles, des familles sont accompagnées de mineurs, contrairement à ce qui se passe dans les CRA. La Cimade dresse un portrait de ces zones : « Être enfermé en zone d’attente, c’est être confronté quasiment tous les jours aux situations suivantes : ne pas pouvoir se soigner, ne pas manger à sa faim, dormir dans des locaux insalubres ou aux conditions d’hygiène dégradées. Allonger ainsi le délai du jugement des requêtes aux fins de maintien en zone d’attente, alors qu’il s’agit d’un enfermement administratif, prive les requérants de leur chance d’être libérés dans les délais les plus brefs. Il s’agit d’une énième atteinte à la dignité et aux droits des personnes migrantes. Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

quelle qu’elle soit, soit justifiée dans son fondement et dans sa nécessité par rapport au but légitime visé et à sa proportionnalité. C’est d’autant plus important lorsqu’il s’agit de personnes qui ne sont ni condamnées ni soupçonnées d’avoir commis un délit ou un crime. Or cet article vise à permettre au juge des libertés et de la détention de statuer dans un délai de quarante huit heures lorsque le nombre d’étrangers placés simultanément en zone d’attente est trop important. Autrement dit, ce texte fait peser sur l’étranger privé de liberté le manque des moyens humains et matériels de la justice. Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article.

Si Mayotte est bien un département français, il n’y a aucune raison que ce système d’exception perdure ! Les conditions de vie sur l’île deviennent insupportables,

de Mayotte, qui a déjà très bien expliqué la situation. Nous ne pouvons pas continuer à contraindre à rester sur le territoire mahorais des mineurs qui sont en situation régulière : ils doivent être autorisés à circuler sur l’ensemble du territoire français.

Monsieur le ministre,

qui viennent à Mayotte, alors, bien sûr, il faudra mettre fin à ce qui est appelé le visa Balladur. Mais il ne serait pas raisonnable pour la République française dans son ensemble et pour Mayotte en particulier de permettre cette libre circulation aujourd’hui.

Je ne veux pas allonger inutilement nos débats, mais je pense que ce que vivent nos compatriotes mahorais mérite que nous nous y attardions. Il faut entendre le cri du cœur de M. le sénateur.

rectifié est retiré. Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles du projet de loi. Je vous rappelle que les explications de vote